doit permettre aux pays de l'Union européenne de relancer leurs économies, gravement touchées par la pandémie. Cette initiative, exceptionnelle par son ampleur, a une signification profonde

Ils ne veulent pas de mutualisation ni de solidarité, seulement des prêts remboursables, alors même que leur situation économique n'est guère plus florissante que la nôtre et qu'ils dépendent très largement des exportations. des exportations. D'ici au prochain Conseil européen, les négociations pour les convaincre de se ranger derrière un plan de relance réellement solidaire La Commission européenne, l'Allemagne, la France doivent les persuader de participer à ce plan, et il reste de nombreux problèmes à résoudre quant aux clés de répartition, aux secteurs concernés, aux modalités de remboursement.

engager la relance économique de l'ensemble des pays européens, confrontés à la crise économique la plus grave de leur histoire, et ce sur la base d'un plan de relance verte. Ce plan reprend l'intégralité des propositions avancées par la Chancelière Angela Merkel et le Président de la République ; cela doit être un motif de fierté pour nous tous.

par l'accord conclu entre les ministres des finances le 9 avril dernier, soit, au total, un plan de relance verte de 1 300 milliards d'euros pour l'ensemble des pays européens. C'est une proposition majeure, qui montre que l'Union européenne est au rendez-vous de l'histoire.

cela aidera tous les États européens à financer leur propre relance, l'investissement dans l'innovation et les nouvelles technologies. J'appelle donc tous les États européens, sans exception, y compris les quatre « frugaux », à soutenir ce plan de la Commission européenne

et tout doit être mis en oeuvre pour qu'elle aboutisse. Elle est nécessaire pour l'Europe, car, soyons honnêtes, le plan de relance de la Commission européenne, dont une partie est fondée

d'autant que la décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe sur la légalité de la politique monétaire de la Banque centrale européenne avait jeté un grand froid. Je rappelle que cette décision remet en cause la solidarité des dettes par le biais monétaire. Le choix franco-allemand d'une approche budgétaire pour soutenir les pays endettés pourrait marquer un tournant. Ce plan traduit-il la solidarité tant attendue par les États membres les plus fragilisés par les conséquences économiques de la crise du Covid-19 ? Ouvre-t-il enfin la voie à la mutualisation des dettes, que Berlin avait toujours refusée jusque-là ? Est-il une réponse à la décision de la Cour constitutionnelle allemande, qui aurait pu affaiblir la politique économique européenne et mettre en péril la zone euro ? Très bien

est historique et marque une avancée majeure dans l'affirmation de l'Union européenne sur la scène internationale, d'abord par l'ampleur des sommes mises sur la table

est à l'origine. Je pense que nous sommes tous ici convaincus que le moteur de l'Union européenne, qui permet de faire avancer les choses, de casser les plafonds de verre, de progresser dans l'intégration européenne, et donc de nous protéger

parce que, pour la première fois, nous acceptons une mutualisation des dettes sur un projet de financement de dépenses budgétaires. C'est intéressant financièrement, parce que cela permet d'obtenir le taux d'intérêt le plus faible possible

à ceux qui ont été le plus touchés par la crise du coronavirus ; oui, nous allons donner plus à l'Espagne et à l'Italie. Ce devrait être un motif de fierté pour nous tous, parce que cela signifie que nous savons aider les États les plus en difficulté. Oui, les États rembourseront

Cette décision aurait été prise lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale. Le choix de cette instance tient sans doute à la nature des manifestations qui se déroulent dans ce parc ; je pense par exemple aux combats de gladiateurs Nous sommes très heureux que l'État, depuis son sommet, donne ainsi la possibilité de retravailler aux nombreux professionnels de la culture du Puy du Fou. Notre peine est en revanche immense pour les artistes, les intermittents du spectacle, les auteurs, les compositeurs, tous ces professionnels sur lesquels repose le rayonnement culturel de notre pays, qui se sentent totalement abandonnés,

Avec eux, ce sont des milliers de structures culturelles qui risquent de disparaître. Tout ce réseau patiemment construit pendant des décennies a fait de notre pays la première destination touristique mondiale. Son activité économique mobilise 2,4 % de la population active et près de 50 milliards d'euros. Il a fait de la culture un service public et donné à nos concitoyens les moyens de leur élévation artistique et de leur émancipation intellectuelle. Ce réseau, d'une grande fragilité, risque aujourd'hui d'être emporté par la crise, alors que nous aurions tellement besoin de culture pour la surmonter. Il ne se passe pas une semaine sans que votre gouvernement n'annonce des plans de sauvetage de plusieurs milliards d'euros. La culture doit, elle, se contenter de proclamations lyriques et de vaines promesses. Monsieur le ministre, à quand un plan de sauvetage de la culture ?

a fait en sorte que les mesures transversales annoncées par le ministre de l'économie et des finances, sous l'autorité du Premier ministre, puissent être accessibles à ce secteur : fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, exonérations de charges sociales,

pris un ensemble de mesures, à la fois d'urgence et d'accompagnement à la reprise, pour protéger ce secteur si durement touché. La

La crise sanitaire que nous traversons entraîne dans son sillage une crise sociale et économique sans précédent. Si le mécanisme de chômage partiel a jusque-là servi de filet social à la crise économique, votre décision de le diminuer, conjuguée au durcissement de l'accès à l'indemnisation imposé par la réforme de l'assurance chômage entrée partiellement en vigueur à la fin de 2019, laisse craindre une précarisation grandissante de nombreux travailleurs. Les travailleurs les plus fragiles, ceux qui, avant la crise, occupaient un emploi précaire, et les travailleurs des secteurs le plus sévèrement touchés par la crise sanitaire, déjà durement affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19, le seront davantage encore avec la réforme de l'assurance chômage. Je pense notamment aux extras de la restauration,

le deuxième volet de la réforme de l'indemnisation du chômage n'est donc pas suffisante, car c'est l'ensemble de la réforme qui pose problème et qu'il faut définitivement abroger. Madame la ministre, la seule volonté qui sous-tend cette réforme est d'atteindre un double objectif comptable, en réalisant des économies budgétaires au détriment de l'indemnisation des chômeurs et en agissant artificiellement à la baisse sur les statistiques du chômage. C'est cette même logique comptable qui a conduit l'hôpital public à la situation alarmante que nous connaissons. Eu égard à l'ampleur de la crise, cette réforme, comme celle des retraites, doit être abandonnée.

Actuellement, le FCTVA est versé deux ans après la réalisation de la dépense aux collectivités territoriales n'ayant pas conventionné avec l'État au titre du plan de relance. Pour celles qui ont

nombreuses sont les communes qui ne disposent pas d'une trésorerie suffisante pour assurer le financement de certains investissements. Aussi doivent-elles contracter des prêts relais qui leur permettront en particulier de couvrir les dépenses de TVA, d'où un coût supplémentaire pour ces collectivités. Cela constitue un véritable frein à l'initiative locale et s'avère pénalisant, dans la mesure où les élus risquent, à long terme, de s'interdire tout projet de développement des équipements locaux, ce qui entraînera une dévitalisation, notamment dans les campagnes. il apparaît indispensable de préserver la capacité financière de nos communes, afin qu'elles soient en mesure non seulement de continuer d'assurer les services essentiels à la population, mais également de relancer les investissements indispensables au soutien au tissu économique local. Afin d'atténuer le choc financier subi par les collectivités locales, les modalités relatives au versement du FCTVA pourraient être modifiées pour permettre une récupération de la TVA dès la première année, notamment pour les communes ayant effectué un investissement

des comptes publics. Monsieur le sénateur, vous avez raison, les collectivités locales sont celles qui investissent le plus et soutiennent l'économie sur l'ensemble du territoire.

ou encore la course à l'échalote à laquelle l'État s'est livré pour se fournir en masques et en médicaments, mettant ainsi à nu notre dépendance sanitaire. Les pays producteurs se servent les premiers, c'est ainsi, et le coronavirus nous l'a rappelé parfois avec cruauté. Des voix se sont élevées pour dire que plus rien ne sera jamais comme avant, selon une formule rituelle et quasiment liturgique. Cela étant, monsieur le ministre, il y a un domaine dans lequel notre pays a gardé une réelle capacité à produire : l'agriculture et l'agroalimentaire. Bien que mal considérés et souvent mal rémunérés, nos agriculteurs assurent notre indépendance alimentaire, et ce en dépit d'une concurrence déloyale qui nous fait perdre du terrain année après année. Comme si les erreurs du passé n'avaient pas servi, la Commission européenne vient à la fois de proposer de réduire de 10 % la superficie des terres cultivables en Europe, et donc en France, et de conclure, après le CETA, un accord de libre-échange avec le Mexique, qui concerne précisément les produits agricoles.

Le combat contre la Covid-19 serait plus efficace avec une meilleure connaissance de la diffusion du virus sur le territoire et de l'intensité de l'épidémie selon les régions. À cet À cet égard, un avis de l'Académie des technologies publié le 19 avril dernier attire l'attention sur les renseignements que peuvent fournir les eaux usées. la mesure de la concentration du génome du virus dans les eaux usées pourrait permettre de mieux évaluer le nombre de malades dans une zone donnée, car le suivi prend en compte les virus rejetés par la totalité des personnes porteuses, qu'elles soient saines, asymptomatiques ou malades. L'information récoltée permettrait aux collectivités locales et aux agences régionales de santé (ARS) d'évaluer avec plus de précision l'état sanitaire du territoire dont elles ont la responsabilité et d'apporter une réponse adaptée. En outre, le coût de telles mesures de suivi serait relativement modeste. Des mesures de surveillance des eaux usées ont déjà été annoncées à l'étranger. En France, le Comité analyse, recherche et expertise (CARE) mis en place par le Président de la République a apporté son soutien à une telle pratique.

Elle a été intégrée à celle de notre collègue Cédric Perrin, déposée voilà plusieurs semaines et adoptée ce matin par la commission des lois. Ce texte a deux ambitions : adapter les opérations de vote à un contexte épidémique persistant et faciliter l'établissement des procurations. Adapter les opérations de vote, c'est garantir aux électeurs qu'ils pourront exercer leur droit de vote sans risque pour eux-mêmes ni pour leurs proches. C'est aussi permettre aux candidats, à leurs représentants et aux membres des bureaux de vote de participer au déroulement et au dépouillement du scrutin en toute sécurité. Je ne sollicite ici aucune faveur ; je demande seulement la considération élémentaire que la République doit à ses citoyens. Faciliter l'établissement des procurations, c'est permettre à chaque électeur de détenir deux procurations, de voter pour un de ses parents proches dans une autre commune que celle où il réside. C'est aussi donner à une personne fragile, âgée, isolée ou malade la possibilité d'établir une procuration à son domicile. Là encore, il ne s'agit que de respecter l'équité républicaine. Il n'y a pas de société démocratique sans vote citoyen. Le freiner ou le tronquer serait un sacrilège. Après l'abstention et les frustrations du premier tour, ce second tour est attendu depuis de nombreuses semaines. Nous devons, vous devez permettre la participation du plus grand nombre d'électeurs. Nous devons, vous devez faire la loi qui le garantira. loi qui le garantira. Nous avons tout mis en oeuvre pour adopter en moins d'une semaine les textes sur l'état d'urgence sanitaire et sa prorogation. Le Gouvernement est-il prêt à utiliser tous les moyens constitutionnels à sa disposition pour faire aboutir ces mesures électorales indispensables avant le 15 juin, afin qu'elles puissent être mises en oeuvre dans de bonnes conditions le 28 juin

de la fracture numérique, qui pénalise lourdement les enfants des milieux modestes, les emplois aidés seraient bien utiles à ceux qui ne savent pas maîtriser un outil devenu indispensable. Étant donné les besoins existants dans les écoles et les collèges et la nécessité de donner un avenir aux jeunes de ces quartiers, le Gouvernement compte-t-il réactiver les contrats aidés ?

un « effet de ciseaux » cruel, entre échéances à court terme et manque de trésorerie pour redémarrer la machine économique post-confinement. De plus, les demandes excéderont les capacités de traitement des banques. Il faudra donc bien diversifier l'offre. européens d'investissement de long terme (Eltif) peuvent souscrire des prêts émis par des plateformes dans le dispositif des prêts garantis par l'État. Les personnes morales ont été exclues de cette possibilité, alors qu'elles ne sont pas moins averties que les personnes physiques et les fonds Eltif. Dans la filière agroalimentaire, en particulier, des groupes de la grande distribution ou de la coopération agricole se sont portés volontaires pour ce type de financements auprès de certains de leurs partenaires habituels. L'intérêt de les intégrer paraît donc évident. Pour éviter des faillites en cascade, il pourrait être utile d'élargir le dispositif de la garantie de l'État aux entreprises qui financeraient une partie du prêt, des plateformes, à des entreprises de leur filière qu'elles connaissent parfaitement.

Monsieur le ministre, j'entends votre réponse. J'avais d'ailleurs salué l'adoption par le Sénat, la nuit du 22 avril, de l'amendement du Gouvernement tendant à intégrer les plateformes de financement participatif de type au dispositif des prêts garantis par l'État.

faire face à la crise actuelle, toutes les forces comptent pour relancer l'économie. Les entreprises qui prêtent à leurs partenaires au sein de leur filière- j'ai fait référence à la filière agricole -ne comprennent pas pourquoi elles ne pourraient pas bénéficier aussi de garanties de l'État, ou de l'Europe

J'informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ont été publiées.

La crise du Covid-19 : révélateur de la dimension cruciale du numérique dans notre société. Quels enseignements et quelles actions ? » Dans le débat, la parole est

Pour certains, il est devenu essentiel, tandis que d'autres l'ignorent ou le tiennent à distance. Nous l'utilisons sans forcément bien comprendre ce qu'il y a derrière, comment tout cela fonctionne. Nous subissons les débordements et les excès des réseaux sociaux, parfois avec un certain fatalisme. Pourtant, nous en voulons toujours plus : plus d'appareils connectés, plus de débit, plus de services en ligne ... La crise du Covid-19 a fait exploser les besoins. Le numérique est devenu l'outil quotidien, du télétravail aux leçons des enfants en passant par les courses en ligne ou la visite virtuelle aux grands-parents confinés. Le confinement a mis en évidence notre extraordinaire dépendance au numérique, toujours plus présent, toujours plus nécessaire, toujours plus demandé ... Nous avons pris conscience de ses formidables potentialités pour rompre l'isolement, maintenir le lien et poursuivre les activités, mais aussi de notre vulnérabilité de notre souveraineté par des réseaux pilotés de l'étranger, qui ne nous garantissent plus la confidentialité de nos données personnelles. Nous avons regretté, une fois de plus, notre incapacité à faire émerger des champions du numérique, nous conduisant à renoncer à notre souveraineté alors que les Français se ruaient en masse vers des solutions américaines. Nous avons pris conscience de l'insoutenabilité d'une fracture muée en gouffre numérique, qui laisse de côté près de 13 millions de nos concitoyens, exclus par choix, par appréhension ou faute de connexion. L'intérêt et les enjeux stratégiques du numérique sont désormais évidents et devant nous. L'accélération des investissements dans les infrastructures, la formation, la recherche sera une priorité incontournable pour le prochain plan de relance. C'est pourquoi que le groupe Union Centriste a souhaité ce débat. d'identifier les carences et les « trous dans la raquette » apparus de manière flagrante pendant cette crise : maillage territorial insuffisant, numérisation des entreprises balbutiante, illectronisme excluant 13 millions de Français, cybersécurité insuffisamment prise au sérieux, protection des données personnelles encore aléatoire, assujettissement à quelques géants mondiaux peu solidaires, manque de compétences et de formation aux métiers, faiblesse des fonds alloués aux start-up, absence de grands industriels capables de soutenir la recherche, de promouvoir la dynamique d'intelligence artificielle et les investissements qui vont avec Fondamentalement, ce débat est d'abord un échange sur la société numérique que nous voulons pour demain, au regard de ce que nous pouvons observer tout autour de la planète, où se dessinent différents types de sociétés du numérique. Les discussions sur l'application StopCovid qui suivront ce débat nous amènent à nous interroger devrons-nous choisir entre sécurité et libertés individuelles ? Sommes-nous prêts à accepter un traçage numérique de notre quotidien et à livrer des données personnelles pour une plus-value sanitaire qui reste d'ailleurs à démontrer, au vu des conditions de sa mise en oeuvre ? Définir le numérique de demain impose donc de mener une réflexion de fond sur le cadre pertinent- national ou européen ? -, sur les engagements financiers et industriels pour s'équiper, sur le soutien massif à l'innovation pour s'adapter, sur les valeurs et l'éthique de régulation qui commencent à émerger avec le européen ou Tech for Good France, réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs acteurs d'une transition durable et responsable. Cette nécessaire régulation doit encore être approfondie, s'agissant notamment des plateformes structurantes et des places de marché. Le Sénat a d'ailleurs déjà fait des propositions en matière d'interopérabilité. Dans un monde numérique sans frontières physiques, dont certains se jouent avec des lois à portée extraterritoriale, comme le américain, bâtir un modèle de société numérique axé sur son utilité et ses externalités, tant sociales qu'environnementales, réfléchir sur le rôle et l'usage de l'innovation sont, on le voit bien, autant de jalons essentiels, reposant en partie sur une politique de la donnée et du partage entre acteurs économiques qui reste encore à construire. Peut-être pourrons-nous alors gagner la bataille des données stratégiques, après avoir perdu celle des données personnelles Dans ce monde numérique où l'intelligence artificielle fait aujourd'hui sa révolution quantique, on parle 5G et nanotechnologies, on réfléchit, tandis que bon nombre de Français peinent à manipuler leur tablette, voire s'effraient de toutes ces perspectives.

Ni les cybercafés, ni les cyberespaces, ni les pass numériques et autres n'ont réussi à raccrocher les 13 millions de Français exclus du numérique. La méthode employée n'était peut-être pas la bonne, monsieur le ministre. Par exemple, le Parlement n'a pas été associé à l'élaboration du mobile en 2018. C'est pourtant ensemble,

société numérique ? La société du gigabit pour 2025 promue par la Commission européenne est-elle aujourd'hui une utopie ? Comment pensez-vous favoriser la numérisation des entreprises françaises, aujourd'hui parmi les plus mal loties d'Europe, notamment après la disparition du fournisseur d'accès Kosc ? Pensez-vous mobiliser les fonds privés en faveur des entreprises du numérique, créer un crédit d'impôt à la numérisation des TPE et des PME, renforcer le suramortissement ?

Le virage du numérique exige la confiance dans le numérique. Trop souvent, nous le voyons, le numérique effraie. Les derniers débats liés à la 5G et à l'utilisation du numérique dans la crise sanitaire en témoignent. Plus concrètement, la recrudescence de la cybermalveillance et des cyberattaques atteste de risques et de menaces bien réels.

Les questions sont nombreuses ; mes collègues y reviendront certainement. Les enjeux liés au numérique sont immenses. Ils fondent, nous l'avons vu, beaucoup de craintes, mais aussi d'énormes espoirs. Cette terrible crise du Covid-19 peut être l'occasion d'une prise de conscience salvatrice de l'impérieuse nécessité de créer une société numérique inclusive et sécurisée

Certains prétendent même que, à terme, grâce au numérique, cette période de confinement pourrait changer les aspirations et les modes de vie des Français, beaucoup d'urbains s'installant dans les territoires ruraux, comme semble l'indiquer la profession immobilière, qui croule sous la demande. Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que, dans cette Haute Assemblée des territoires, on imagine aussi un numérique pouvant changer le destin des territoires, transformer le visage de la France et faire renaître des provinces jusque-là délaissées ! La parole

Essor du télétravail, enseignement à distance, émergence de la télémédecine, traçage de la transmission du virus : la crise du Covid-19 a donné une place encore plus importante au numérique dans notre quotidien. Au fil des jours, notre pays s'est transformé en véritable start-up internet, le taux de connexion, durant ces derniers mois, ayant atteint des niveaux largement supérieurs à ceux constatés l'année dernière à la même époque. Bien entendu, une telle tendance se faisait déjà jour au sein des entreprises, dans les pratiques domestiques ou encore au sein des services de l'État. S'agissant en particulier de l'administration, elle a accéléré sa mue depuis quelques années, avec la dématérialisation croissante des démarches administratives.

souscrire. Cependant, il y a des obstacles à franchir, le principal étant de permettre à tous nos concitoyens d'accéder à internet et d'avoir un minimum d'aptitudes numériques. En lorsque la transition numérique en laisse un certain nombre au bord de la route ou pose question quant au respect des libertés publiques, c'est notre pacte républicain qui est abimé.

L'inclusion numérique, c'est l'autre grand défi à relever pour réussir la transition. Si la période de confinement a permis d'enrichir les compétences numériques de beaucoup de nos concitoyens, elle a pu aussi fragiliser encore un peu plus les familles en situation de précarité. À l'école, assurer la continuité pédagogique par le biais d'internet était sans doute la seule option pour permettre au plus grand nombre d'enfants possible de continuer à suivre les cours, mais les dégâts pourraient être irréversibles pour ceux qui n'ont pu s'inclure dans le système. Bien sûr, là aussi, la crise du Covid-19 n'a fait que souligner un phénomène connu, qui mobilise déjà les pouvoirs publics. J'en profite pour rappeler le travail réalisé par le Sénat à travers la mission d'information sur la lutte contre l'illectronisme et pour l'inclusion numérique que le groupe RDSE a souhaité mettre en place pour apporter des réponses à l'exclusion numérique. En tant que président de la Commission supérieure du numérique et des postes, je voudrais souligner l'action de la Banque postale, qui conduit un programme national d'accompagnement des publics en difficulté à travers 300 bureaux de poste. Par ailleurs, beaucoup de collectivités locales mettent en oeuvre des stratégies d'inclusion, avec la création de tiers lieux dédiés aux usages numériques. Malgré cette mobilisation, il reste d'importants efforts à mener pour réduire cette fracture sociale. Cela pourrait passer par un développement des aides à l'achat d'équipements informatiques, par davantage de soutien à la formation numérique gratuite, ainsi que par une simplification des applications pour les démarches publiques. Enfin, mes chers collègues, une autre conséquence inattendue de l'épidémie, c'est l'accélération de l'entrée de la santé dans le monde numérique. Sur ce point, je n'évoquerai qu'un seul enjeu, celui des libertés publiques, qui est au coeur des débats sur l'application StopCovid. Nous aurons l'occasion d'en reparler ce soir, mais je rappellerai ici les précautions qui doivent entourer l'usage d'une application numérique de traçage. Le retour à la libre circulation des citoyens et la reprise économique sont des priorités

liberté du consentement des usagers et citoyens, anonymat des usagers et des données collectées, respect des règles de proportionnalité, sécurité renforcée des technologies employées, caractère provisoire du dispositif, caractère ouvert, c'est-à-dire auditable, de la technologie employée. Mes chers collègues,

ce débat ambitieux sur l'importance cruciale du numérique dans notre société à l'heure de la crise du Covid-19. Répondre en quelques minutes, de manière pertinente et panoramique, à cette vaste et complexe question relève

à ce stade de la crise, ou plutôt des crises provoquées par la pandémie du Covid-19, de tirer aujourd'hui des enseignements sinon définitifs, tout au moins objectivement et quantitativement évaluables, de l'impact de cet événement dans tous les domaines de la société aujourd'hui pénétrés par la numérisation. Bien sûr, le roi n'est pas nu, et nous disposons de quelques données sur des aspects aussi importants que le recours significatif au télétravail par les entreprises et les salariés au plus fort du confinement, l'usage accru des grandes plateformes de distribution de services et de produits, tant physiques que dématérialisés, la progression singulièrement forte des enseignements à distance dans le domaine de l'éducation et de la formation, l'usage prononcé du numérique en substitution à la consommation en physique et en présentiel de l'information, du divertissement et de la culture ... Que sais-je encore ? Mais ces données nous permettent-elles de savoir si nous sommes véritablement à un tournant de la numérisation de la société ? Sont-elles prédictives, secteur par secteur, de ce que seront les usages et les pratiques à venir, ou sont-elles

de vivre, ou va-t-on progressivement revenir à une tendance antérieure à la numérisation de la société, observée bien avant la crise du Covid-19 ? La réponse à ces questions n'est pas simple. Je prendrai deux exemples pour illustrer mon propos : ceux du livre numérique

transformé l'industrie phonographique, en France comme à l'étranger. La dématérialisation a également transformé l'industrie cinématographique, celle du jeu vidéo ou encore la presse écrite et l'information en général. Ce que l'on note, concernant le livre numérique, c'est que, après un début de décollage, il y a une quinzaine d'années, il n'y a pas eu par la suite de véritable

Pourtant, à l'occasion du confinement et de la fermeture des librairies et des bibliothèques au public, nous avons assisté à un engouement nouveau pour le livre numérique. Que va-t-il se passer à présent ? Depuis leur réouverture, les librairies semblent retrouver leur clientèle, et c'est une bonne chose. Les lecteurs semblent encore très attachés au livre physique, par nature délinéarisable, annotable, exhibable, donnable, prêtable ou échangeable Pour autant, nombre de librairies indépendantes, de petits et de moyens éditeurs sont aujourd'hui dans une situation économique des plus précaires. S'ils disparaissent, que deviendront la lecture ainsi que le livre et ses modes de diffusion classiques ? L'offre numérique ne risque-t-elle pas de prendre économiquement le dessus sur le livre physique, et la distribution par l'entremise des grandes plateformes numériques ne va-t-elle pas menacer les plateformes physiques et les librairies ?

risque d'une « activité zéro » qui aurait ruiné notre économie. Nous avons, à cette occasion, découvert des ressources nouvelles que nos entreprises comme leurs salariés n'imaginaient pas auparavant.

Le télétravail a ses avantages et ses bénéfices, mais aussi ses défauts et ses coûts. Gardons-nous surtout d'en théoriser les bienfaits ou les méfaits- hors période de peur généralisée de la pandémie -avant d'avoir étudié de manière plus approfondie ce qui s'est passé

sera indispensable de fonder un nouveau contrat social ou, en tout cas, un nouveau contrat de travail entre employeurs et salariés, afin que ces derniers ne soient pas les dindons de la farce d'une telle

que, à l'aune de la crise actuelle, nous entrons peut-être dans une troisième phase de la relation des citoyens au numérique et à internet. La première phase, ce fut la période des débuts, la période utopique où internet symbolisait

L'accès à internet sur l'ensemble du territoire est devenu un véritable droit prioritaire pour chacun. Une enquête de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir de l'an dernier nous apprend que 6,8 millions de personnes, soit 10 % de la population française,

On observe dès lors une fracture entre deux mondes, chacun vivant à la vitesse de ses capacités de connexion : les métropoles branchées d'un côté, la France profonde, enracinée mais déconnectée, voire oubliée, À cette fracture numérique s'ajoute la crise sanitaire actuelle. Elle révèle les promesses, les insuffisances et les dérives du numérique. Le numérique a permis aux familles séparées de se voir, au monde du travail de poursuivre son activité à distance et en sécurité, à nos commissions parlementaires de continuer à se réunir. Avec le télétravail, les entreprises ont adopté de nouvelles habitudes pour l'avenir.

une solution de facilité pour sortir du confinement. C'est une dérive. Il y a également la menace que fait peser le télétravail sur nos libertés, par la remise en cause des conditions de travail. Il y a un risque de glissement, sur lequel il faut rester vigilant. Le fameux « métro-boulot-dodo » ne doit pas devenir « boulot-boulot-boulot Une mauvaise séparation entre vie privée et vie professionnelle pourrait conduire à une multiplication des risques psychosociaux. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : le télétravail ne doit pas devenir la règle imposée ; il doit garder son caractère exceptionnel et relever d'un choix personnel. Le télétravail doit rester une nouvelle possibilité de flexibilité ponctuelle pour les travailleurs. J'ai entamé mon propos en évoquant une révolution du numérique : nous le savons, toute révolution produit des excès. Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour que le numérique prenne sa place, toute sa place, mais rien que sa place dans notre société ? Le numérique doit rester un moyen : le havre de paix de la vie privée doit être sacralisé.

où le droit à la mobilité et la liberté d'aller et venir se sont trouvés restreints. Comment continuer à apprendre, à comprendre, à travailler alors que l'on est assigné à résidence ? Les fractures et les inégalités se sont indéniablement trouvées renforcées.

des pistes d'action. Tout d'abord, il est clair que le numérique, ou plutôt l'accès au numérique, est apparu pour ce qu'il est : un pan essentiel du service public de la communication et de l'information. Pour cette raison, nous demandons, malheureusement sans succès jusqu'à présent, l'intégration du très haut débit au service universel. Nous espérons que, à la lumière de cette expérience, la définition du service universel pourra évoluer. L'ensemble de nos concitoyens doivent pouvoir accéder au numérique. C'est un droit qui conditionne l'accès à l'enseignement, au travail, à la santé, aux loisirs, à la culture et à l'information. Pourtant, aujourd'hui, les progrès restent trop faibles en matière de raccordement, puisque près de 15 % du territoire est mal couvert. Les objectifs définis par les opérateurs sont rarement respectés, faute de véritables sanctions. Les collectivités territoriales, qui assument une part majeure de l'investissement dans les réseaux d'initiative locale, ne sont pas suffisamment soutenues.

L'investissement public a, une nouvelle fois, été détourné au profit d'actionnaires, à contresens de l'intérêt général. Cela devrait nous interpeller et nous conduire à placer sous protection publique les réseaux à très haut débit, dont l'accès est si important pour nos concitoyens. Toutes les infrastructures de communication, qu'elles soient routières, aériennes ou numériques, doivent être sous maîtrise publique ; cela comprend les aéroports, les autoroutes, mais aussi la fibre. Cette crise doit également nous amener à nous interroger sur nos modèles d'aménagement urbain. Le logement, structure de base de l'habitat, mais aussi, et de plus en plus, du travail, ne peut plus être à ce point le parent pauvre des politiques publiques. Puisque les liens sont plus plus forts que les lieux, la structure première qu'est le logement doit redevenir une priorité des politiques publiques, au même titre que l'enseignement. Sur ce sujet, nous avons pu voir comment le numérique a renforcé les fractures à l'école. Lors de l'annonce de la fermeture des établissements d'enseignement, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal ont promu la « continuité pédagogique ». Deux mois et demi plus tard, on ne peut que voir les failles d'une telle démarche. En voulant En voulant simplement transposer l'enseignement de la classe à la maison par le biais de l'ordinateur, sans donner les outils nécessaires aux enseignants, l'éducation nationale n'a fait que creuser les inégalités entre les élèves inégalités d'accès aux outils informatiques et à un débit convenable, inégalités de maîtrise des outils et du travail en autonomie, inégalités d'environnement de travail et d'accompagnement. Le retour à l'école n'a pas profité aux jeunes en difficulté, alors que c'était l'objectif affiché.

Le numérique, indispensable outil d'apprentissage à l'école lorsqu'il s'appuie sur un véritable encadrement pédagogique, ne pourra remplacer ni la présence dans les établissements scolaires ni l'apprentissage de la vie sociale et collective. Il serait dangereux d'utiliser cette crise pour déshumaniser le service public de l'enseignement. l'un des faits les plus marquants de cette crise est la généralisation du télétravail. La violence de l'épidémie a entraîné une évolution immédiate des méthodes de travail pour des milliers de salariés, de travailleurs indépendants et de professionnels libéraux. Rappelons toutefois

et rapidement déchanté au vu des conditions imposées depuis le 16 mars. La permanence du télétravail, la nécessité de garder les enfants, l'impréparation en termes de formation et de matériel ont parfois transformé cet épisode de travail à la maison en un cauchemar. Comme l'indiquait un expert dans un article récent, « les salariés parlent d'abandon, de solitude, de surcharge cognitive liée au trop grand nombre d'informations à traiter, de surcharge de travail, d'un sentiment d'être surveillé à l'excès par les managers, des difficultés à coopérer avec les collègues et de l'impossibilité de concilier vie privée et vie professionnelle ». D'ailleurs, de nombreux cas de détresse psychologique sont recensés. Les salariés confrontés à des difficultés de transport et au stress de la vie urbaine aspirent à passer moins de temps au travail. Dans cet objectif, le télétravail doit être organisé dans le respect des droits et selon des plages horaires précises, avec des remparts contre le harcèlement numérique. Mais ne faut-il pas se dégager de cette problématique

Le 5 mars dernier, Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne chargée du numérique, appelait à faire des choix clairs pour notre futur. La crise que nous traversons exacerbe la nécessité de penser la place du numérique dans la société non pas demain, mais dès aujourd'hui. Le numérique n'est pas entré dans nos vies en mars 2020, mais il est devenu incontournable dans plusieurs pans de notre société et de notre quotidien. Le Parlement doit s'emparer de ce sujet majeur, car, si les avancées sont notoires, les limites le sont tout autant, et une adaptation de notre système est primordiale.

Je souhaite saluer le travail impressionnant fourni par la majorité du corps professoral pour s'adapter, durant la crise et encore aujourd'hui, et réorganiser la vie scolaire. Ce travail, parfois bien compliqué, a permis à notre jeunesse d'avoir accès à l'enseignement à distance, et ce fut un succès dans beaucoup de cas. Cependant, comme nombre d'entre nous, j'ai aussi noté des limites, et même des fractures profondes dans notre société.

ou, dans le pire des cas, lorsqu'aucun accès n'est possible. Tous les enfants n'ont pas les mêmes besoins en matière d'éducation. Les parents ne peuvent pas encadrer les enfants comme le font les professeurs, dont c'est le métier. Tous les élèves ne disposent pas d'un espace suffisant pour se concentrer et suivre de manière assidue un enseignement en ligne.

Cependant, l'enseignement ne peut pas se faire uniquement à distance et des supports numériques. L'humain doit rester au centre de la transmission. Les deux approches, loin d'être incompatibles, doivent être appréhendées comme complémentaires. L'enseignement à distance peut être très utile, par exemple pour les enfants malades, qui peuvent

Depuis mars, notre regard sur le sujet a évolué et chacun a pris conscience des avantages que le télétravail pouvait apporter aux entreprises et aux salariés, si bien que, des grandes entreprises aux start-up, les adaptations ont été rapides et de nouvelles organisations

par semaine à domicile, il devient intéressant de s'installer à une heure d'une métropole. Enfin, les entreprises y trouvent aussi leur intérêt, en réduisant les coûts grâce à une réorganisation des locaux. beaucoup de questions se posent ; je n'en évoquerai que quelques-unes : l'isolement social de la personne en télétravail, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le volet juridique du télétravail ou encore l'accès à internet. Toutes ces interrogations nous incitent à envisager un système hybride, donnant sa juste place au numérique. Je voudrais rappeler qu'environ 20 % des Français n'ont pas accès à internet ou sont reliés à un réseau de mauvaise qualité. Il reste encore des citoyens vivant en zone blanche, même si des progrès sont à l'oeuvre. accéder au numérique est vraiment essentiel, son absence étant synonyme de difficultés et d'isolement. Le numérique est donc bien crucial dans notre société. De nombreuses facettes positives ont été dévoilées. Il reste maintenant à mener une large réflexion, au regard tant de la place

Ses usages n'ont cessé de se diversifier pour répondre aux différents besoins des Français : le recours au télétravail s'est massifié, la téléconsultation s'est répandue, l'enseignement à distance s'est généralisé. Autant de changements nécessaires, mais adoptés dans la précipitation du fait de la pandémie. Alors que le déconfinement est bien engagé, il paraît approprié de dresser un premier bilan des évolutions radicales qu'ont connues les Français dans leur rapport au numérique durant ces derniers mois. Pour ma part, si je crois cette démarche essentielle, je crains toutefois qu'elle n'occulte la priorité en la matière, à savoir résorber la fracture numérique pour que tous les Français soient égaux devant ce qui devrait relever du service public. Cette carence a généré un nouveau fléau, l'illectronisme. Malheureusement, ce phénomène n'est pas marginal, puisque, selon le Défenseur des droits, un quart de la population française n'a toujours pas accès à internet ou ne sait pas utiliser les outils numériques. De même, dans 75 % de nos communes de moins de 1 000 habitants, la couverture par le réseau n'est pas suffisante pour équiper 100 % des foyers. Ce n'est pas acceptable Le plan France Très haut débit vise à corriger partiellement cette situation, par la couverture de 80 % du territoire d'ici à 2022, mais la crise sanitaire va causer de nombreux retards, empêchant de tenir cet objectif. Dans ce contexte, je tiens à saluer l'ordonnance

Quant aux territoires ruraux, des plans pour la couverture en très haut débit sont mis en oeuvre dans de nombreux départements, avec des projets de déploiement de la fibre optique jusqu'à l'habitation. Pour des raisons économiques, la desserte par la fibre des zones rurales ne s'opèrera pas en souterrain, mais en aérien, en utilisant les lignes des réseaux préexistants. Or on constate,

À mon sens, cela limiterait le retard du déploiement de la fibre dans le monde rural et permettrait à ce dernier de connaître les changements sociétaux suscités par le numérique. Monsieur le ministre, le Gouvernement a dit que le numérique serait un pilier de la relance économique, mais comment comptez-vous accompagner concrètement les différents acteurs de la filière, privés comme publics, de manière que tous les Français puissent avoir accès au numérique dans des conditions optimales ? La parole

Quel bilan doit-on tirer de ce test ? La réponse n'est pas univoque. Côté pile, les moyens de communication numérique se sont affirmés, pour la première fois à grande échelle, comme de formidables outils de résilience et de garantie de la continuité de pans essentiels de la vie de notre nation. Les réseaux ont tenu, alors qu'au début du confinement on pouvait légitimement craindre des engorgements, voire des saturations. Cela n'a pas été le cas, et nous pouvons nous en réjouir. Côté face, la crise sanitaire a révélé les failles et les injustices de notre société numérique. Des millions de Français ont ainsi subi une double peine : en plus du confinement, beaucoup ont connu un isolement numérique intolérable, les coupant parfois de leur travail, de l'éducation, de la santé et de leurs proches. La fracture est double. Certains sont déconnectés faute de compétences numériques ou de terminaux pour communiquer- on parle alors d'illectronisme -, d'autres n'ont pas accès à des réseaux fixes ou mobiles de qualité. Ainsi, plusieurs milliers de zones blanches mobiles doivent encore être résorbées. Près de la moitié du territoire n'est pas couvert en très haut débit fixe. Pis encore, une connexion en « bon » haut débit, permettant de réaliser des recherches internet de base, est encore attendue par des milliers de nos concitoyens, alors que le Gouvernement a promis un accès à ce « bon » haut débit pour tous les Français d'ici à la fin de l'année. Il revient aux pouvoirs publics de gagner la bataille de l'aménagement numérique du territoire, au travers des programmes France Très haut débit pour le fixe et New Deal pour le mobile. Le premier vise une couverture intégrale du territoire en très haut débit en fixe pour 2022 et en fibre optique pour 2025. Le second a notamment pour ambition de faire basculer l'ensemble des antennes mobiles existantes en 4G d'ici à la fin de l'année et de résorber des milliers de zones blanches d'ici à 2025, par le déploiement d'un dispositif de couverture ciblée. Malheureusement, la crise sanitaire menace la tenue de ces objectifs. On peut certes se féliciter que certains chantiers aient pu se poursuivre pendant la période de confinement, quand d'autres secteurs étaient à l'arrêt- je voudrais, à cet instant, saluer les acteurs de la filière. Il est cependant probable que certaines échéances ne pourront pas être tenues. C'est ce qui ressort des auditions que j'ai menées pendant le confinement pour la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable avec mes collègues Guillaume Chevrollier et Jean-Michel Houllegatte. Il faut Il faut tirer plusieurs leçons de ces constats. Premier enseignement, la crise ne doit pas empêcher le régulateur- l'Arcep -d'exercer son pouvoir de contrôle et de sanction en cas de non-respect des objectifs assignés aux opérateurs, en adaptant, s'il le faut, les échéances au contexte. Une chose est certaine : il faudra étudier les demandes de report des échéances formulées par les opérateurs au cas par cas et ne pas accepter n'importe quel retard justifié par la crise, d'autant plus que des doutes avaient été émis, avant même le début du confinement, sur le respect de certaines échéances, tant pour le fixe que pour le mobile.

La crise sanitaire démontre pourtant par les faits l'incroyable effet de levier des réseaux numériques sur les activités économiques et la modestie d'un tel investissement au regard de ses effets positifs. Il est certain que l'épidémie du Covid-19 impliquera des surcoûts pour les programmes de déploiement. La rallonge de 322 millions d'euros votée par le Sénat en décembre dernier et rejetée par le Gouvernement ne serait donc peut-être plus suffisante

Je suis convaincu que nous pouvons, sur certains sujets techniques, trouver de nouveaux leviers de simplification. Nous devons aussi accélérer le déploiement de la base adresse nationale. Aujourd'hui, 30 % des foyers français ne sont pas couverts par la base adresse, ce qui occasionne des difficultés de raccordement à la fibre. Ce taux est encore plus fort dans les territoires ruraux. Nous devons remédier à cela, par exemple en donnant très clairement la compétence aux maires pour la dénomination des voies et l'adressage et en confiant à l'Agence nationale de la cohésion des territoires la responsabilité d'accompagner les collectivités territoriales dans l'élaboration de leur base adresse locale.

les faire avancer. La parole est à Mme Viviane Artigalas. La crise sans précédent que nous traversons a bouleversé nos usages et nos habitudes de vie. Ces deux mois de confinement, d'autant plus difficiles à vivre que la situation était inédite, ont été rendus en grande partie supportables grâce au numérique. À la faveur de la crise, l'accès de tous au numérique est apparu comme un nouveau droit fondamental, celui de bénéficier, quel que soit le territoire, d'une connexion internet suffisamment opérationnelle pour pouvoir travailler, se soigner et accéder aux services publics dans de bonnes conditions.

La fracture numérique soulève la question centrale de l'inclusion des territoires et des usagers. J'ai déjà alerté le Gouvernement sur le sentiment d'abandon et d'insécurité ressenti par les habitants des territoires ruraux et montagnards. La crise a clairement illustré les inégalités territoriales en matière de numérique. Certains cumulent les handicaps en termes de réseau, de matériel, de capacités d'utilisation. Mon collègue Jean-Michel Houllegatte complètera mon propos, qui est centré sur l'inclusion numérique. numérique. La fracture numérique peut, chez nos concitoyens, se manifester par un manque de maîtrise des usages et des outils du web, que ce soit à cause de l'âge, du niveau de formation, d'un handicap ou, tout simplement, de difficultés de lecture. Monsieur ainsi évalué à 13 millions le nombre de Français qui ne savent pas se servir d'internet ; 20 % de la population a ainsi un accès limité ou inexistant aux procédures dématérialisées.

Pôle emploi, agences de l'habitat ... -plaçait déjà nombre de nos concitoyens dans une situation de grande fragilité technologique. Si la dématérialisation peut permettre une simplification et un gain de temps, elle doit être accessible à tous, ce qui n'est pas le cas actuellement. En effet, elle s'est parfois faite dans l'urgence et de manière radicale, sans aucune préparation, sans formation ni accompagnement à l'usage des nouveaux outils, qui sont complexes. Cela limite l'accès aux aides de l'État pour certains de nos concitoyens, particulièrement les plus fragiles. Ces difficultés concernent également les entreprises, notamment les plus petites d'entre elles- je pense par exemple à la dématérialisation des marchés publics. Or ces difficultés d'accès aux services publics mettent à mal l'égalité républicaine, et la crise a considérablement accentué ce phénomène. C'est d'autant plus dommageable qu'internet est un outil de résilience qui peut nous aider à relancer l'économie et à améliorer le quotidien de nos concitoyens. Si l'accès au numérique devient un droit fondamental pour tous les Français, il faut que l'État le garantisse au même titre que le droit à un logement digne ou la liberté d'expression. Cela passe par la reconnaissance d'un véritable service public de la médiation numérique et le déploiement de moyens massifs pour accompagner les publics les plus éloignés du numérique. Nous formulons à ce titre plusieurs propositions, dont je ne citerai que les principales conditionner l'objectif de 100 % des services publics dématérialisés en 2022 à la couverture numérique complète du territoire et à l'inclusion numérique ; coconstruire les plateformes numériques avec les usagers faire en sorte que l'inclusion numérique passe nécessairement par l'échelon local, en créant un maillage de médiation numérique qui s'appuiera sur les communes ; mettre en place un accompagnement personnalisé d'ultraproximité qui permette d'aller vers les exclus du numérique équiper chaque foyer d'un matériel informatique performant d'ici à 2022 et optimiser le recyclage des équipements informatiques obsolètes enfin, pour servir ces quelques objectifs, redéployer le fonds pour la société numérique de la Caisse des dépôts et consignations, qui représente tout de même 4,5 milliards d'euros. Le numérique a un rôle capital à jouer pour contribuer à forger une société plus égalitaire, sobre et durable. La sortie de crise ne pourra faire l'économie d'une nouvelle stratégie en matière numérique, et nous savons tous à quel point nous n'avons pas le droit de manquer ce tournant, sauf à prendre le risque que nos droits fondamentaux,

Or la fracture numérique que nous connaissons n'est pas seulement technologique et liée à l'insuffisante couverture du territoire en haut débit ; elle est également culturelle. Rechercher des informations, accéder à ses comptes en ligne, consommer, communiquer mobilise désormais des ressources nouvelles et la maîtrise des outils et langages numériques. Dès lors, la formation au numérique n'est pas une option, la lutte contre l'illectronisme doit devenir une grande cause nationale. C'est le constat que la mission d'information sur l'illectronisme, que j'ai l'honneur de présider, a dressé dès le début de ses travaux, en tirant les leçons de cette terrible épidémie qui a désorganisé nos vies et anesthésié notre économie. Il y a urgence à lutter contre la fracture numérique. L'administration se dématérialise à très grande vitesse. Il y a vingt ans, 4 500 contribuables seulement déclaraient leurs revenus en ligne, contre plus de 20 millions de foyers en 2017.

et qui avait alerté, dès avril 2018, sur les conséquences d'une dématérialisation trop rapide des services publics. Une minorité significative de la population française ne maîtrisant pas le numérique risque de voir ses droits reculer. Pour prévenir une telle situation et réussir l'inclusion numérique, tout doit être fait pour embarquer le plus grand nombre. Il faut d'abord des financements à la hauteur des enjeux, et donc importants. À côté des 20 milliards d'euros du plan France Très haut débit, les financements publics alloués à la résorption de l'illectronisme de 13 millions de Français éloignés du numérique sont-ils à la hauteur ? Il faut ensuite une mobilisation de tous les acteurs, soutenue par une volonté politique forte, évitant une dispersion et concentrant les énergies. L'inclusion numérique est l'affaire de tous. Dans ce domaine, l'État intervient, comme souvent, de manière sans doute trop dispersée

Une coconstruction de stratégies locales est souhaitable pour lutter efficacement contre l'illectronisme. L'école doit apprendre aux élèves à comprendre la Toile dès le collège. Elle doit construire l'égalité des savoirs numériques, notamment au regard des genres, alors que le numérique exprime trop souvent une suprématie masculine. Il faut enfin que l'illectronisme soit pris en considération dans toutes les politiques publiques de manière transversale. Pour éduquer nos concitoyens au numérique, l'école doit approfondir les apprentissages des usages du numérique. Pour les salariés, la formation professionnelle devra intégrer cette dimension. Pour mettre en oeuvre leurs actions, les administrations doivent prendre en compte la non-maîtrise du numérique. Déployer des infrastructures, dématérialiser les procédures, enrichir sans cesse les plateformes de e-commerce de nouveaux produits et services : ce monde d'après que nous préparons doit tenir compte de l'illectronisme. Ayons l'ambition collective d'éradiquer celui-ci, afin de ne pas laisser un trop grand nombre

de nos concitoyens et de nos entreprises. À cet égard, j'admire la réactivité des entreprises, qui, quelle que soit leur taille, se sont adaptées au choc du confinement et à l'arrêt brutal d'activité. Nous avons tous des exemples, dans nos territoires, d'initiatives prises dans les entreprises pour trouver des solutions ingénieuses, adapter leur production, la commercialisation, leurs modes de travail et de management. Production de matériels sanitaires, vente par internet,,, télétravail, visioconférences : la créativité et l'agilité des Français ont trouvé à s'exprimer. Le Sénat se bat depuis longtemps pour l'accès à la fibre pour tous, et la délégation aux entreprises du Sénat travaille depuis près de dix-huit mois sur la question cruciale de la numérisation des entreprises, en particulier des PME et TPE.

la délégation aux entreprises du Sénat a montré que, malgré le succès de ses start-up, la France se caractérise par le retard pris par les TPE et PME pour opérer leur transformation numérique : le classement européen DESI place la France au quinzième rang en 2019.

pérenniser le dispositif de suramortissement pour les investissements de robotisation et de transformation numérique des PME-TPE et permettre l'inscription à l'actif du bilan de l'ensemble des investissements matériels ou immatériels concernés donner à l'Arcep les moyens d'agir avec réactivité pour contrôler le respect des engagements pris par les opérateurs de télécommunications et prendre éventuellement des sanctions ; renforcer l'efficacité de l'Autorité de la concurrence en transposant dans les meilleurs délais la directive ECN+ du 11 décembre 2018. nous avons souhaité aller plus loin. C'est pourquoi j'ai proposé à notre collègue Patrick Chaize, président du groupe numérique du Sénat, de mener des travaux conjoints dès l'automne 2019. Ils ont donné lieu à un rapport d'information, adopté en décembre dernier, dont le titre est révélateur : « Accès des PME à la fibre : non-assistance à concurrence en danger ? ». En effet, au-delà des services de télécommunications, les services numériques et les innovations associées doivent demeurer compétitifs. Pour cela, deux éléments sont essentiels : l'accès au très haut débit et l'accompagnement de l'écosystème numérique. perspective, les opérateurs doivent avoir accès au réseau FTTH, afin de pouvoir offrir des conditions économiquement viables pour les PME-TPE en développant une concurrence effective et loyale sur le marché de gros des télécommunications d'entreprise. Or, malgré la volonté des pouvoirs publics, les résultats ne sont pas à la hauteur. Nous déplorons aussi que les PME soient les victimes de défaillances en matière de complétude. Ce retard provient largement d'un manque de dynamisme de l'écosystème des services numériques aux entreprises, dû notamment aux restrictions dans le dégroupage des infrastructures fibre pour le marché des télécommunications d'entreprise par rapport au marché résidentiel. La concurrence par ce dégroupage existe en effet seulement dans les zones « réseau d'initiative publique » (RIP), où les entreprises bénéficient d'un meilleur niveau de services, à des conditions tarifaires favorables. Dans les autres parties du territoire, la régulation de la concurrence sur le marché des télécommunications d'entreprise doit être améliorée afin de favoriser une réelle concurrence sur le marché de la fibre à destination des TPE et PME. Ainsi, nous défendons l'« intérêt général numérique », sujet sur lequel nous alertons le Gouvernement depuis près d'un an. C'est pourquoi nous déposerons dans quelques jours, avec Patrick Chaize, une proposition de loi en ce sens. Elle visera à renforcer la concertation entre les deux autorités de régulation et à conforter la finalisation de l'ouverture à la concurrence du marché des télécommunications d'entreprise par la régulation. Ce sujet technique recouvre des enjeux stratégiques majeurs pour l'adaptation de nos PME aux défis d'aujourd'hui. Nous n'avons plus d'autre choix que d'agir vite pour soutenir nos entreprises et leurs salariés, où qu'ils soient. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour soutenir notre démarche. La parole

de notre société, un bien essentiel, un nouveau droit, un service de base, au même titre que l'eau et l'électricité. Aussi devons-nous saisir l'occasion de la transcription en droit français de la directive européenne concernant le service numérique universel pour engager un débat au Parlement, afin de définir les contours et les modalités Les réseaux ont tenu face à l'accroissement significatif des usages : le trafic internet a en effet augmenté de 20 % à 30 % et le trafic voix a été multiplié par Mais la crise a mis aussi en relief les fragilités liées aux fractures numériques, qu'elles soient territoriales ou sociales, comme l'a souligné avant moi Viviane Artigalas. Les naufragés du Net,

Concernant la fracture territoriale, nous devons poursuivre et accélérer le déploiement des réseaux, dont le rythme s'est ralenti. Certes, les opérateurs, hormis la fermeture des boutiques commercialisant produits et services, ont été peu impactés, à l'inverse des entreprises de BTP ou de maintenance, qu'il faut continuer à soutenir, sauf à perdre les compétences durement acquises ces derniers temps, qui ont permis à la filière de livrer 4 millions de prises en 2019. Les réseaux d'initiative publique, qui démontrent chaque jour que les infrastructures sont un bien commun, doivent être soutenus par le biais du guichet numérique afin de boucler les plans de financement.

Enfin, concernant la téléphonie mobile, les engagements du New Deal doivent être tenus. Mais cette crise a aussi mis en relief la vulnérabilité du Net et, sans doute, la nécessité de nouvelles régulations. La ruée vers le numérique a fait que les noms d'applications comme Webinaire, Zoom ou BlueJeans sont passés dans le langage commun. Dans la précipitation, nous avons produit de la donnée, entrouvert les portes de nos systèmes d'information, alors que la cybercriminalité individuelle ou organisée, y compris étatique, n'a cessé de progresser. Nous devons, au plan national, renforcer notre action pour la production de services numériques sécurisés

La régulation doit concerner également les flux, pour éviter les embouteillages sur les nouvelles autoroutes de l'information. D'ailleurs, les opérateurs ont appelé les consommateurs à faire preuve de « civisme numérique Même si les principaux acteurs, comme Netflix, ont réduit de 25 % l'intensité de trafic et si YouTube a paramétré ses vidéos, par défaut, sur une qualité d'image standard, voire dégradée, la crise met en évidence le poids considérable pris par le vidéo dans les usages numériques : il représente environ 50 % du trafic internet en France ! Elle met aussi en lumière notre dépendance aux grands acteurs du, presque tous américains, et nous incite à revisiter, certes avec précaution, le principe de neutralité du web pour canaliser les flux liés à ces usages vidéo.

Monsieur le ministre, cette crise démontre la nécessité de construire une stratégie numérique républicaine englobant les infrastructures, les services et les usages, pour un numérique durable au service de tous nos concitoyens.

La crise confirme malheureusement la pertinence des positions défendues par notre commission et notre assemblée depuis tant d'années. « Malheureusement », car on ne peut pas se réjouir d'avoir raison, alors que confinement a rimé avec isolement pour des millions de Français éloignés du travail, de l'éducation, de la santé, faute d'un accès satisfaisant aux infrastructures numériques. J'appelle donc le Gouvernement à prendre acte de ces constats et à placer l'aménagement numérique du territoire en bonne position dans les priorités Je m'exprime également en tant que corapporteur de la mission d'information relative à l'empreinte environnementale du numérique, lancée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en janvier dernier. Je rappelle que le numérique représente environ 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Ce chiffre pourrait doubler d'ici à 2025. La croissance de l'empreinte environnementale du numérique est extrêmement inquiétante

Je considère que le numérique ne continuera à être un facteur de continuité des activités essentielles de notre nation qu'à condition d'être plus sobre. Cela devra être une exigence de la relance. Il ne fait pas de doute que, dans nos territoires, les projets « », comme les projets de ville intelligente, vont se développer. Ces projets visent parfois à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à diminuer la pollution urbaine en fluidifiant le trafic. Il convient de systématiser les évaluations environnementales préalables à ces opérations de numérisation, en intégrant notamment une analyse du cycle de vie des équipements numériques installés. Pour cela, il faut donner aux acteurs les moyens de quantifier les impacts environnementaux associés à certains usages et à certains équipements. Notre mission d'information préconisera de mettre à disposition du public une base de données afin de permettre aux entreprises et aux administrations d'évaluer les incidences environnementales de leurs programmes de numérisation. L'information environnementale doit également être disponible pour les consommateurs. À titre d'exemple, nous avons parfois observé, pendant le confinement, un report de la connexion à l'internet vers les réseaux mobiles, pourtant beaucoup plus énergivores et fragiles que les réseaux fixes. Dans certains cas, les réseaux mobiles sont trop largement sollicités les smartphones, malgré la disponibilité des réseaux fixes. Il existe donc des pratiques non optimales, qui menacent la résilience des réseaux et dégradent le bilan environnemental du numérique. Nous sommes convaincus qu'une meilleure information du consommateur sur l'impact environnemental de sa connexion mobile est nécessaire. Dans certaines zones, en revanche, le report vers les réseaux mobiles démontre l'insuffisant déploiement de la fibre : on se connecte son smartphone à la 3G ou à la 4G faute de mieux.

de nombreux concitoyens en ont fait l'expérience pendant le confinement. Nous devons donc aujourd'hui tendre vers une plus grande sobriété des services numériques. Plusieurs pistes sont d'ores et déjà étudiées par la mission d'information. Ainsi, le lancement automatique de vidéos, qui ralentit considérablement le chargement de certaines pages, pourrait être

Voilà quelques premières pistes que notre mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique a explorées. Nous ne manquerons pas, monsieur le ministre, de vous détailler dans les semaines et les mois à venir les résultats de nos travaux. Une chose est certaine : nous avons aujourd'hui l'occasion de bâtir une société numérique

M. le ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord m'associer aux nombreux remerciements qui ont été adressés

Un tel débat ne peut, bien entendu, laisser de côté la crise actuelle, mais nous voulons le rendre plus aigu, en interrogeant la mondialisation telle que nous la connaissons et telle que nous la souhaitons. En tant qu'Européens convaincus, nous avons la chance de pouvoir influer sur le cours de cette mondialisation, même si beaucoup en doutent, au premier rang desquels les Européens eux-mêmes.

la question légitime qui se pose : comment faire en sorte que la France et, plus largement, l'Union européenne s'assurent une indépendance stratégique, notamment en matière sanitaire ? Dans un premier temps, il nous faut comprendre les ressorts de la localisation des entreprises.

En réalité, les délocalisations nous ont permis d'accéder à des marchés émergents à croissance rapide tout en faisant baisser nos coûts. À titre d'exemple, seuls 4 % des investissements directs français correspondent à des délocalisations motivées par des différences de coûts salariaux et impliquant la réimportation des produits finaux. Néanmoins, le mouvement de délocalisation conduit à des spécialisations régionales qui font émerger un modèle économique opposant les activités de conception, dans les pays du Nord, à celles de production, dans les pays du Sud. La crise actuelle a démontré qu'une telle situation

justifiées par des problèmes de qualité des produits, des augmentations des coûts de personnel ou encore des coûts de coordination et de suivi. Souhaitons-nous, dès lors, envisager une nouvelle vague de relocalisations ? Si le constat semble unanime, quels en seraient alors les ressorts ?

telles aides risquent surtout d'attirer des chasseurs de primes, ces entreprises nomades ou volatiles qui quittent le territoire à l'approche de la fin de la période d'exonération. En réalité, les relocalisations pérennes s'expliquent par des motifs de compétitivité par l'innovation, et non par les prix. si nous souhaitons relocaliser une partie des productions stratégiques, privilégions donc les relocalisations néo-schumpetériennes d'innovation plutôt que les relocalisations tayloriennes visant à une baisse des coûts. Je pense, bien sûr, à la recherche médicale, mais également à l'hydrogène en tant qu'énergie de rupture technologique propre non seulement à conforter notre souveraineté, mais également à nous donner une avance technologique. Dans un second temps, il nous faut comprendre les limites des relocalisations et définir des ambitions industrielles renouvelées. Depuis les années 1990, les investisseurs américains comme européens se sont plutôt tournés vers la semi-périphérie asiatique que vers le voisinage proche ; il nous faut en partie inverser la tendance. Ne confondons pas pour autant vision stratégique et discours souverainiste ! Ce dernier fait le constat que la souveraineté économique ne coïncide plus avec la souveraineté politique. diagnostic lucide, quoique tardif, d'une fragmentation des chaînes de valeur, mais prôner un retour en arrière s'opérant uniquement sous les injonctions d'un État-nation fantasmé est totalement vain. Face à la régionalisation caractérisant actuellement la mondialisation, nous avons une chance à saisir : celle d'une souveraineté industrielle européenne.

permettent aux États membres de soutenir des projets transnationaux d'importance stratégique, qu'il s'agisse de la microélectronique ou, plus récemment, des batteries électriques. nous exemptons pas pour autant d'une réflexion nationale sur notre industrie, que nous devons impérativement moderniser ! À ce titre, l'industrie du futur constitue une occasion unique de rendre l'industrie française plus attractive et compétitive. Si la France possède des atouts pour accélérer son déploiement, les efforts à cette fin doivent être rationalisés au regard de la trop grande fragmentation des dispositifs de financement, d'accompagnement et de formation. Que l'on veuille produire sur notre sol des produits de première nécessité, quand c'est indispensable, ou surtout des produits stratégiques à forte valeur ajoutée, la question des coûts de production et de la nécessaire baisse de la fiscalité de production

revient au politique de lui donner un sens afin de relativiser les bienfaits de la main invisible smithienne. La relocalisation des productions stratégiques passe alors par l'identification des secteurs essentiels à notre pays, ainsi que par des mesures que par des mesures ciblant les défaillances spécifiques du marché, comme l'illustre l'impérative nécessité de faire de tout vaccin un bien public mondial.

Si nous refusons le confort idéologique consistant à prôner un protectionnisme aveugle et vain, nous appelons en revanche de nos voeux une souveraineté européenne renouvelée et l'esquisse d'une Europe de la santé,

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il aura fallu une pandémie sans précédent pour que l'organisation industrielle mondiale soit ouvertement contestée. La crise sanitaire que nous vivons a remis sur le devant de la scène la question de la localisation des processus de production des biens considérés comme stratégiques.

Il nous faut produire davantage sur notre sol pour réduire notre dépendance. La forte demande de masques, de respirateurs ou de certains médicaments nous a conduits à nous interroger sur la localisation de certaines productions que l'on juge devoir absolument faire revenir sur notre territoire, pour des raisons d'indépendance et de souveraineté. L'industrie pharmaceutique s'est plus que jamais révélée être un secteur stratégique pour permettre aux États de protéger leur population en cas de besoin. Comme nous le savons tous, la mondialisation a engendré une fragmentation croissante des chaînes de valeur à travers le monde, en permettant que chaque élément de ces chaînes soit fabriqué dans le pays où les avantages comparatifs sont les plus importants. Cette logique a conduit nos pays industrialisés à se concentrer sur la production de biens et services à haute valeur ajoutée, à se spécialiser dans le haut de gamme. Nos coûts de production étant deux fois plus élevés que ceux des pays émergents, les délocalisations ont permis de réduire de 15 % à 20 % le prix du bien industriel consommé en France. Dans les pays riches, où les compétences sont disponibles, mais les salaires élevés, la relocalisation exigerait une forte automatisation de la production, ne créerait pas beaucoup d'emplois et pourrait faire baisser le pouvoir d'achat. concernant la production de médicaments, la France jouit d'un excédent commercial extérieur de taille envers les pays émergents. Nous continuons de gagner des parts de marchés, alors que nous importons la majeure partie des principes actifs basiques, comme le paracétamol, dont la production ne nécessite pas un niveau élevé de qualification des ingénieurs. que jamais, l'opinion publique souhaite un retour massif de la production industrielle sur le sol national. Mes chers collègues, je crains que la crise ne nous amène à imaginer de fausses bonnes mesures. Je ne crois pas à l'idée selon laquelle un certain nombre de productions à faible valeur ajoutée, mais considérées comme stratégiques, devraient être relocalisées. La France n'a pas vocation à relocaliser la production de principes actifs basiques ou de masques. Comment pourrait-on produire à des prix décents des principes actifs à faible valeur ajoutée ? ? Relocaliser ce type de production n'est pas la bonne stratégie. L'industrie pharmaceutique française doit se concentrer sur les produits biotechnologiques les plus innovants. Mes chers collègues, le manque de masque durant la crise est lié non pas à notre dépendance à l'égard des pays étrangers, mais plutôt au manque de stocks en France. La France doit non pas relocaliser ses productions industrielles, mais se réindustrialiser. La nuance est de taille ! L'effort de réindustrialisation doit porter sur des biens à haute valeur ajoutée et s'inscrire dans un agenda européen. Nous savons d'ailleurs que la France est en retard pour le développement des industries de demain

Tout d'abord, parler de souveraineté sans parler des traités européens qui empêchent le patriotisme économique, cela manque d'honnêteté. Aujourd'hui, l'État ne peut pas défendre nos entreprises, car le droit communautaire l'en empêche. C'est l'Union européenne qui a ouvert la porte à la désindustrialisation de notre pays et à l'exode de nos fleurons vers les pays émergents. Nous avons été les grands naïfs de la mondialisation malheureuse, et nous le sommes encore ! Avant de parler de relocaliser, il faudrait déjà penser à protéger les quelques entreprises qui survivent encore chez nous et à les soutenir. La souveraineté économique de la France n'est possible que si nous engageons avec détermination un bras de fer avec la Commission de Bruxelles. Si nous avons manqué de masques, de gel et de tests, c'est parce que nous avions eu l'aplomb de penser- par idéologie ! -que nous pouvions nous passer de notre industrie. Les dirigeants politiques ont appris à leurs dépens- ce n'est pourtant pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme ! -que l'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. La loi du marché ne fait pas de cadeau : les Américains nous l'ont rappelé en rachetant un stock de masques qui nous était destiné sur le tarmac d'un aéroport chinois. toutes les industries, tous les savoir-faire, puissent s'implanter ou se réimplanter dans notre pays. Dans cette perspective, nous ne pouvons nous contenter des propos contradictoires de l'exécutif. D'un côté, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, déclare que « notre objectif est la souveraineté économique de la France le Premier ministre, Édouard Philippe, affirme quant à lui que l'Union européenne n'a pas « été à la hauteur de la crise ». De l'autre, le président Macron vit toujours dans le monde des idées. Il a toujours plus d'ambitions, mais pour l'Union européenne qui importe à ses yeux, ce n'est pas l'intérêt de notre économie, mais le fait que le « manque de solidarité pendant la pandémie risque d'alimenter la colère populiste » ... On le voit, ses intérêts sont idéologiques et électoralistes ! De plus, il faut une réforme fiscale profonde, notamment de l'impôt de production, qui est actuellement le plus élevé en Europe, encourager les entreprises à rester en France. Il faut soutenir les entreprises en continuant de les accompagner par des dispositifs de chômage partiel, car c'est maintenant qu'elles vont subir les conséquences de la crise sanitaire. Il est enfin urgent d'alléger les charges qui pèsent sur elles.

La souveraineté ne peut être que nationale, elle ne saurait être diluée ! Là où la mondialisation ultralibérale soumet à l'interdépendance, le localisme et la souveraineté procurent la liberté : liberté face aux puissances, liberté face au marché, autonomie en cas de crise. En février, au Parlement européen, la droite de M. Bellamy et les marcheurs de Mme Loiseau ont voté main dans la main un accord de libre-échange avec le Vietnam. Rien n'a changé, malgré les promesses de la campagne des Relocaliser les productions stratégiques exige de la cohérence, mais la classe politique continue à croupir dans les eaux usées du libre-échange forcené.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis trente ans, nous constatons la désindustrialisation de la France. En quinze ans, nous avons perdu plus d'un demi-million d'emplois industriels petite musique : cette évolution était inéluctable, la faute à la compétition internationale et à ce que vous appelez « le coût du travail ». D'autres faisaient l'éloge de la déréglementation, de la dérégulation et de la privatisation des entreprises et des monopoles publics.

Pour vous, la partition était jouée d'avance. Le capitalisme financiarisé avait gagné et la fin de l'histoire était actée. Chaque pays devait se spécialiser à raison de ses avantages comparatifs, puis échanger

l'accaparement des richesses et des profits par la minorité qui détient le capital. Chaque fois que nous osions remettre en question ce système, on nous riait au nez. Lorsque nous parlions nationalisation ou monopoles d'État, souveraineté coopérante ou projets industriels, nous n'étions pas entendus.

Pour vous, tout doit être marché, tout doit être profit, tout doit être précaire, comme le disait la patronne du Medef il y a quelques années. Pour rivaliser avec les autres pays, vous nous répétiez qu'il n'y avait qu'une solution casser le code du travail, allonger la durée du temps de travail, faire sauter le SMIC, étouffer les syndicats, bloquer les salaires, faire travailler les salariés plus longtemps et, surtout, aider les entreprises. Et les salariés ! Des aides, beaucoup d'aides, trop d'aides : crédit d'impôt pour la

cette crise a révélé nos insuffisances. Nous ne savons plus produire certains biens, y compris des biens de première nécessité. Imaginons un seul instant notre réaction si l'on nous avait dit, il y a seulement quelques semaines, que, dans la sixième puissance mondiale, des équipes soignantes seraient réduites à découper des sacs poubelles pour s'en servir en guise de surblouses ... Oui, la « start-up nation »a montré son incapacité à protéger les Français ! Alors que des questions se posent à nouveau avec force, nous voulons prendre toute notre place dans ce débat. Nous proposons un autre chemin : il s'agit de s'appuyer sur la relocalisation et la nationalisation de pans entiers des secteurs stratégiques, afin d'amorcer la nécessaire transition écologique

en même temps un plan de restructuration faisant planer une sérieuse menace sur sa filiale Hop ? Trouverons-nous normal de prêter 5 milliards d'euros à Renault sans prise de participation dans cette entreprise, qui laisse planer une menace de fermeture sur quatre usines représentant 3 200 emplois,

mettons-nous d'accord : il est urgent de revenir sur l'autorisation administrative de licenciement en période de crise, mesure qui n'a jamais créé les centaines de milliers d'emplois annoncés. Il est aussi urgent de revenir sur les décrets Macron de 2017 pour aboutir à une conception plus protectrice des licenciements économiques. Nous vous proposons ensuite de prolonger d'urgence le dispositif de chômage partiel pour tous les secteurs jusqu'au 31 décembre et de soumettre les aides et les prêts garantis par l'État à des critères sociaux et environnementaux. Les prêts aux grandes entreprises doivent être convertis en montées au capital ou en nationalisations. Ensuite, à court terme, il faudra renforcer le décret Montebourg et étendre la liste des secteurs stratégiques, par exemple au secteur du médicament ou à celui des banques et des assurances, dont on a vu le rôle dans cette crise.

taxe carbone aux frontières européennes -doivent être discutés sereinement entre nous. La crise sanitaire a mis en évidence la nécessité absolue de produire en France du matériel médical et sanitaire. Alors, agissons dès à présent pour construire le pôle public du médicament

deux secteurs nous apparaissent prioritaires : ceux de l'énergie et des transports. Il faut revenir sur la privatisation d'Engie, annuler le projet Hercule, qui vise à scinder EDF en deux entités, réfléchir à la création d'un pôle public de l'énergie qui garantirait un prix à l'usager et amorcer ainsi la transition écologique.

et de réfléchir à un projet industriel du XXI siècle en vue de construire le train du futur, un train plus rapide, plus efficace, plus écologique. Voilà les quelques pistes que nous soumettons au débat : nous allons continuer, avec vous,

Le choc de la crise a obligé tous les pays à réagir très vite, rarement de façon coordonnée, en mobilisant leur système de santé et leur tissu économique. Nul n'était prêt à faire face à ce virus. Tous les gouvernements ont été confrontés à une même réalité : le monde est interdépendant. sont apparues, car le temps est passé où l'État disait et l'administration suivait. Nous n'avons pas renoncé à notre souveraineté ; simplement, les temps ont changé. On ne peut pas construire la souveraineté nationale au XXI siècle comme on le faisait au siècle dernier. Le débat d'aujourd'hui porte sur la relocalisation des productions stratégiques. Je veux commencer mon propos par une clarification : la crise du Covid-19 n'est pas une crise de la mondialisation. La mondialisation n'est pas la cause de la crise ; celle-ci n'en a pas non plus montré les limites. Ne cédons pas aux discours simplistes ! La mondialisation des échanges profite aux producteurs comme aux consommateurs. Ce n'est pas l'interdépendance qui pose problème, mais la seule dépendance. De ce point de vue, la théorie économique et le bon sens paysan convergent : il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Nous ne devons pas jouer l'économie de marché mondialisée contre la souveraineté nationale : la seconde ne s'acquiert que par la première. L'histoire l'a déjà prouvé et le prouvera encore. Pour ceux qui en douteraient encore, il suffit de penser aux deux plus grandes économies mondiales. Les États-Unis comme la Chine ont acquis leur puissance par l'économie de marché et le commerce international. Dans les deux cas, malgré des trajectoires totalement différentes et même opposées, l'ouverture à l'international constitue la clé de la puissance. ces deux exemples nous incitent aussi à ne pas faire preuve de naïveté en matière de souveraineté. Il faut confronter la théorie économique au principe de réalité. Ici encore, les exemples des États-Unis et de la Chine sont révélateurs. D'un côté, la Chine, le plus libre-échangiste des pays communistes, se développe par un capitalisme d'État qui veille surtout aux intérêts nationaux, quitte à verrouiller son marché intérieur.

Dans les deux cas, de grands groupes privés agissent comme les bras armés d'un pouvoir politique. Je ne pense pas que nous devions suivre leur modèle, mais je sais aussi que nous ne devons pas en subir les conséquences. Nos valeurs doivent non pas nous affaiblir, mais nous renforcer. nos entreprises sont l'objet de convoitises étrangères. C'est le cas de nombreux fleurons industriels français. Nous devons faire preuve de lucidité, car un rachat par une entreprise étrangère peut nuire à nos intérêts stratégiques. Je pense au rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric au regard de la maintenance de nos réacteurs nucléaires. Je tirerai de ces exemples trois leçons pour la préservation de nos intérêts stratégiques. D'abord, la souveraineté passe par le maintien sur le territoire national des centres de décision plus que des unités de production. Il faut miser sur les activités à forte valeur ajoutée pour peser sur les décisions stratégiques. Ensuite, pour défendre nos valeurs de liberté et d'innovation, mieux vaut miser sur les forces du marché que sur une économie administrée. C'est dans cette logique que doit s'inscrire notre politique économique. Enfin, pour peser face aux géants, la France a besoin de l'Europe. La révolution numérique a fluidifié les échanges et les communications. Nous devons miser sur notre capital humain et encourager la circulation des talents et des idées à l'échelle européenne. Il s'agit donc d'adapter le projet humaniste qui se trouve au fondement du rêve européen à la réalité du XXI siècle. Cela passe notamment par la révision de nos règles de concurrence, afin de favoriser l'émergence de géants européens. Nous avons besoin de nouveaux groupes du type d'Airbus dans plusieurs secteurs. Mes chers collègues, l'esprit français est toujours tiraillé entre des instincts contraires. Comme nous avons eu Voltaire contre Rousseau, nous avons eu Turgot contre Colbert. L'un et l'autre peuvent nous inspirer Nous avons besoin d'entreprises françaises aussi fortes qu'indépendantes. Cela nous oblige à faire preuve de réalisme et de détermination face aux puissances étrangères prédatrices de nos fleurons industriels. Des solutions existent pour protéger nos entreprises sans que l'État contrôle l'économie. Par exemple, instaurer la taxe carbone aux frontières permettrait à nos entreprises d'être sur un pied d'égalité avec leurs concurrentes étrangères, et ce sans nuire à la dynamique du marché. Notre souveraineté ne passera pas par le recours à une économie administrée. Laissons les énergies s'exprimer dans tous les territoires. Laissons parler Turgot

avec la crise sanitaire, les Français ont pris conscience de la faiblesse de notre industrie, dont ils n'imaginaient pas l'extrême fragilité, entraînant une dépendance de la France dans des secteurs essentiels à notre société. Cette situation concerne le monde

La crise du Covid-19 a agi comme un révélateur de l'urgence de repenser notre organisation, afin de disposer d'outils efficaces pour que la France et, plus largement, l'Union européenne puissent s'assurer une indépendance stratégique industrielle. présent, une vision économique prudente consistait à multiplier les fournisseurs pour ne pas faire dépendre son approvisionnement d'une seule entreprise. Or la crise sanitaire a mis en lumière que, au-delà des fournisseurs, il pouvait être dangereux que l'approvisionnement dépende d'une seule zone géographique. La crise a mis en évidence la nécessité de contrôler certaines activités stratégiques, particulièrement la chaîne de production et d'approvisionnement de matériel médical, de principes actifs, de produits anesthésiants comme le curare. Notre dépendance en la circonstance s'est révélée problématique, dans la mesure où les décisions dû être prises en fonction de la disponibilité des stocks. Notre collègue Catherine Fournier ne dirait pas autre chose ... Dès lors, le principe de souveraineté commande non pas d'étudier la nécessité même de relocaliser certaines productions- elle s'est imposée d'elle-même mais de travailler dès maintenant sur les modalités de la démarche : quelles relocalisations ? Où et comment ? Si la crise sanitaire a servi de catalyseur à l'examen de la question des relocalisations, il faut élargir le spectre, la prochaine crise mondiale ne mobilisera peut-être pas les mêmes productions. En effet, si nous voulons que la réflexion sur la souveraineté ait une réelle portée, il faudra identifier l'ensemble, ou du moins l'essentiel, des « productions stratégiques », lesquelles ne peuvent être circonscrites aux seuls produits médicaux et pharmaceutiques. Il s'agit d'abord des produits de première nécessité, ceux qui sont liés à l'idée que l'on se fait de l'indépendance et de la souveraineté. À ce titre, outre celui des produits médicaux,

fondée sur les productions de première nécessité correspond à une conception défensive des relocalisations et de la souveraineté, nécessaire mais pas suffisante. La stratégie industrielle doit

Il faudra nécessairement prendre en compte, dans l'analyse, tous les diagnostics environnementaux et numériques pour accompagner ces mutations industrielles, que Thierry Breton nous avait présentées lors de son audition devant la commission des affaires économiques

Il faudra répondre à la question : où relocaliser ? La complexité de l'identification des secteurs stratégiques ne pourra être surmontée sans aborder la question de la relocalisation au sein de l'Union européenne : le marché intérieur français ne suffit pas. La crise doit amener un sursaut de l'Union européenne. Celle-ci ne pourra se relancer qu'en élaborant une réflexion sur la production industrielle au sortir de la crise sanitaire. La notion de mondialisation va évoluer. Les attentes des populations vont changer.

Le système multirégional permettra de se rapprocher des marchés de proximité et des lieux de consommation, de réduire l'empreinte carbone des produits et, par là même, d'être plus compétitif. Afin de déterminer où relocaliser les productions stratégiques, il faudra mener une démarche multipartite avec le monde industriel, France Industrie, l'État, en lien avec l'Europe, les régions, les intercommunalités. Madame la secrétaire d'État, comment le Gouvernement entend-il engager ce chantier de la relocalisation industrielle et selon quels modes de coopération avec tous ces acteurs ? Il faudra répondre à la question des moyens à mettre en oeuvre pour faciliter ce tournant industriel. La stratégie industrielle post-crise sanitaire commande que l'Union européenne préserve sa souveraineté, mais aussi maintienne et développe son poids économique avec des outils adéquats. Instaurer la taxation carbone aux frontières de l'Union européenne est une nécessité. Pour restaurer des conditions de concurrence équitables, il faut une politique volontariste de la Commission européenne, qui doit se saisir pleinement de nouveaux outils de défense commerciale, ceux existant aujourd'hui étant insuffisants et peu adaptés. Il faut absolument les réviser, à un rythme différent du européen habituel. Par ailleurs, quels moyens l'État entend-il mettre à disposition des entreprises ? Quel plan d'investissement prévoit-il pour les accompagner dans la mise en oeuvre de leur stratégie de relocalisation ou de réorientation de leur activité économique vers la production de biens à forte valeur ajoutée ? La question des fonds propres se posera avec acuité. La question de la fiscalité de production sera inévitablement posée. Attention aux fausses bonnes idées

des hommes et des femmes de notre pays. Il faudra que l'État engage une simplification des obligations administratives. Il faudra sans doute aussi inventer de nouveaux outils financiers, à l'instar des partenariats public-privé,

l'un des principaux enseignements de cette crise est qu'elle nous rappelle le rôle structurant de l'industrie et sa nécessaire revalorisation dans notre politique économique. La réorientation, voire le tarissement de certains flux de produits industriels, qui ont résulté sont un rappel à l'ordre : il est certains produits, certaines activités dont la Nation ne peut se passer. Le risque est trop grand pour la santé publique, pour l'activité de notre pays ou pour

Bien sûr, nous ne pourrons pas tout relocaliser, tout produire sur notre territoire national. Cela n'est d'ailleurs pas nécessaire ni possible, mais nous devons conduire une réflexion stratégique sur nos priorités industrielles. Il faut en tout cas faire renaître le débat sur une plus grande proximité entre le lieu de production et le consommateur et le consommateur : outre l'enjeu stratégique, c'est également un enjeu environnemental, un enjeu de société, car il y va du lien entre les Français et leurs territoires. Madame la secrétaire d'État, c'est sur ces objectifs et les moyens de cette relocalisation que je souhaite vous interroger.

Vous avez déclaré que la fiscalité doit être l'un des outils de la relocalisation. Quelles pistes étudiez-vous, alors que le pacte productif aurait dû traiter de ce sujet

Parlons de l'Europe. Les règles européennes encadrent strictement les aides que l'État peut dédier à la relocalisation, alors que le Japon offrira près de 2,2 milliards d'euros de subventions aux entreprises rapatriant leur production. Pour que l'Europe ne soit pas de nouveau à la traîne,

plus proche de nous et avec qui nous sommes historiquement, géographiquement, économiquement liés. Très bien ! Il offre tout autant d'opportunités pour sécuriser et diversifier notre approvisionnement. Le Gouvernement entend-il relancer et approfondir cette coopération économique ? Il me semble que c'est un bon moment

Bruno Le Maire a déclaré lundi que vous ne demanderiez pas de contreparties, en termes de relocalisation, à Renault, à qui nous nous apprêtons pourtant à consentir un prêt garanti de 5 milliards d'euros, sur les 8 milliards d'euros du plan automobile. Madame la secrétaire d'État, je pense qu'il ne faut pas reculer.

le Parlement et les partis politiques répondent « présent », car nous n'avons pas le droit de gâcher les enseignements de cette crise.

la crise due au Covid-19 a jeté une lumière crue sur notre dépendance à l'égard d'acteurs lointains. Elle nous invite ainsi à reconsidérer en profondeur notre système économique, avant de le relancer. La France, sixième puissance économique mondiale, qui possédait le meilleur système de santé du monde il y a encore quelques années, s'est pourtant trouvée fort démunie face à cette épidémie. Au nom d'un modèle présenté comme « l'horizon indépassable de l'humanité », notre pays a été progressivement réduit à l'impuissance : système hospitalier et recherche publique affaiblis, tissu industriel démantelé, entreprises et savoir-faire délocalisés Avec la crise engendrée par cette pandémie, on se rend finalement compte que ceux qui ont privilégié une logique de rentabilité immédiate plutôt que de soutenir l'investissement dans les secteurs stratégiques étaient davantage les cigales que les fourmis de la fable. La prise de conscience de la nécessité de retrouver de la souveraineté est désormais largement partagée et transcende certains clivages politiques, comme le démontre le débat aujourd'hui. Au sein du groupe socialiste et républicain, nous avons travaillé, ces dernières semaines, selon une démarche prospective, pour préparer le « monde d'après », et pouvons ainsi apporter quelques réponses aux questions posées à l'occasion de ce débat sur la relocalisation des productions stratégiques. productions ? Les secteurs clés que nous identifions sont la santé, l'alimentation, l'énergie, les transports, le numérique, sans bien sûr oublier les productions industrielles qui se sont révélées indispensables dans la crise. La présence d'entreprises industrielles dans nos territoires conditionne de fait le maintien de nos emplois. Aussi la reconquête industrielle ne doit-elle pas se réaliser au détriment des territoires ruraux. Ceux-ci doivent profiter des plans de relance et de relocalisation industrielle. Comment ? En assumant une rupture claire avec les politiques d'austérité menées ces dernières années et en prenant systématiquement en compte la préoccupation environnementale pour la reconstruction de notre système de production. À la vision idéologique du « tout marché », nous proposons de substituer une vision pragmatique et d'analyser la faisabilité d'une relocalisation secteur par secteur. Plus largement, notre assemblée a déjà produit de nombreuses réponses à ces questions, à travers différents travaux conduits ces dernières années. Mme Létard l'a mentionné : voilà un an, la mission d'information sur l'avenir de la sidérurgie préconisait un engagement fort de l'État pour soutenir cette filière, symbolique du déclin de l'industrie dans notre pays, pallier les défaillances du marché et relever les grands défis, comme celui de la décarbonation. La crise a encore révélé d'autres faillites de notre appareil productif, particulièrement insupportables dans le secteur sanitaire.

particulièrement visionnaire ! Même si elle mettait plutôt l'accent sur le risque de catastrophe climatique, elle nous alertait sur la grande dépendance alimentaire de nos territoires et le ballet de camions qu'elle induit. Le degré d'autonomie alimentaire de nos territoires n'est que de 2 % en moyenne, alors même qu'ils disposent d'actifs agricoles permettant de couvrir 54 % des besoins de leurs habitants. Il ne manque donc que la volonté politique pour organiser la reconnexion entre production et consommation. Dans tous les cas, la relocalisation de nos productions doit s'accompagner d'une reconversion écologique de notre industrie et de notre agriculture. Cela implique, d'une part, un engagement massif de l'État dès le prochain plan de relance, et, d'autre part, un conditionnement des aides d'État à un engagement des entreprises dans la transition écologique, ainsi qu'au maintien de l'emploi et des investissements en France. Bien entendu, la reconversion écologique de notre industrie et la réindustrialisation de nos territoires doivent pouvoir s'appuyer sur l'Union européenne,

qui mettent à mal nos normes protectrices. Enfin, cette reconquête industrielle doit être socialement inclusive, pour que l'on puisse véritablement s'attaquer à l'extrême pauvreté révélée par la crise, mais présente depuis des décennies en raison du creusement des inégalités. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons disposer d'indicateurs autres que le PIB, qui n'est que purement quantitatif et monétaire. Le groupe de réflexion sur les nouveaux indicateurs de richesse, créé sur l'initiative de notre collègue Franck Montaugé, a déjà produit deux propositions de loi particulièrement bienvenues pour penser le « monde d'après De même, nous devons nous emparer de la notion de biens communs, qui questionne les limites de la marchandisation de la nature et du travail. C'est que vient de faire notre collègue Nicole Bonnefoy en déposant une proposition de loi visant à inscrire dans la Constitution les principes de protection du sol et de garantie de la souveraineté alimentaire. Ainsi, les outils et les moyens pour relocaliser nos productions stratégiques ont, pour beaucoup, déjà été pensés sur ces travées. Le Covid-19 et la crise qu'il a induite ont joué un rôle de révélateur de la trop grande dépendance de notre pays dans plusieurs secteurs clés.

collègues, je remercie le groupe Union Centriste d'avoir permis la tenue de ce débat sur un sujet dont la crise du Covid-19 a révélé toute la pertinence. La relocalisation des productions était déjà présente dans le débat avant cette crise sanitaire, mais les récents événements

à penser la construction de notre indépendance dans de nombreux secteurs essentiels à la Nation. Avoir dans cet hémicycle un débat sur la relocalisation des productions stratégiques pour assurer notre souveraineté est fondamental à cet égard. Avant d'évoquer la relocalisation des moyens de production, il convient de s'interroger sur le maintien des outils existants afin de préserver ces outils et d'éviter

380 personnes, dont l'outil de production est neuf et la qualité de production reconnue, ferme au moment même où l'on se soucie de relocalisation et où la puissance publique soutient fortement le groupe Renault par l'apport de gros moyens financiers. Il en est de même pour trois autres filiales de Renault. De manière générale, il convient de réfléchir collectivement aux conditions de la relocalisation. Comment garantir un retour en France des industries sans rentrer dans la course au moins-disant social et environnemental ? Comment garantir l'accessibilité, pour les plus pauvres, des biens produits en France, qui seront qui seront souvent plus coûteux, du fait de normes plus exigeantes ? Relocaliser signifie aussi repenser nos politiques de lutte contre les inégalités. Enfin, je pense que, à plus long terme, la souveraineté ne passe pas uniquement par une relocalisation de la production ou la constitution de stocks stratégiques : elle passe aussi par une réduction de nos besoins, donc de notre dépendance. nous ne pouvons pas nous passer de médicaments, mais combien de maladies pourraient-elles être évitées grâce à une politique de santé axée sur la prévention ? En matière énergétique également, les gisements d'économies sont particulièrement importants. la suite de mon propos au secteur de l'alimentation. S'il est une production stratégique, c'est bien celle-ci. La souveraineté alimentaire des territoires, dont on parle de plus en plus, plus, passe par un certain nombre de ruptures. Même si la France reste une puissance agricole, la vulnérabilité de notre modèle a également été mise en lumière pendant cette crise.

sur le lien entre résilience alimentaire des territoires et sécurité nationale. Les analyses sur les tensions et les risques de rupture d'approvisionnement en cas de crise qui le fondent ont montré toute leur pertinence. que la crise du Covid-19 ne doit en aucun cas être dissociée de l'urgence climatique, qui pèse aussi grandement sur la résilience de notre modèle alimentaire. Relocaliser l'agriculture, ce n'est surtout pas revenir sur nos exigences environnementales pour produire plus. Ce n'est pas poursuivre dans la voie d'un modèle agroindustriel responsable de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre et participant à l'effondrement de la biodiversité, à la déforestation, à la dégradation de la qualité des sols, de l'air, de l'eau. Ce n'est pas poursuivre dans la voie d'un modèle qui, on le sait, détruit des emplois agricoles et la vie dans les territoires ruraux, l'agrandissement sans fin des exploitations ; un modèle qui engendre de la détresse chez celles et ceux qui parviennent, non sans peine, à se maintenir à flot. La transition agricole et alimentaire est attendue par une partie grandissante de notre population ; elle passe à la fois par une relocalisation des productions et par une transition vers l'agroécologie, en vue d'assurer la souveraineté alimentaire de nos territoires. Les solutions sont déjà amorcées localement l'agriculture biologie diversifiée, qui approvisionne les circuits courts, mais de nouvelles filières doivent être organisées sur les territoires pour garantir une autonomie à l'échelle

réussir la souveraineté alimentaire des territoires nécessitera d'augmenter la population agricole et le nombre de fermes, de préserver totalement les terres agricoles, de favoriser l'autonomie technique et énergétique des fermes, de diversifier les variétés cultivées, avec des semences adaptées aux terroirs pour pouvoir affronter les crises qui nous attendent, d'adopter une gestion intégrée de la ressource en eau pour faire face aux menaces de sécheresse, de diversifier les productions pour satisfaire localement aux besoins de la population, de sortir, l'agroécologie, de la dépendance aux pesticides,

Ces principes devraient être appliqués sur l'ensemble de nos territoires, mais aussi sur toute la planète. Cela n'implique bien sûr en aucun cas la fermeture aux échanges, mais ceux-ci doivent se réaliser dans le cadre d'un commerce juste et équitable, respectueux du droit fondamental à l'alimentation des populations, au rebours au rebours de la logique des accords de libre-échange. Pour parvenir à la relocalisation de l'alimentation sur les territoires, un vaste plan est nécessaire, assorti de financements pour accompagner la transition agricole, l'organisation des filières de proximité, ainsi que la généralisation des projets des projets alimentaires territoriaux, outils qui ont fait leurs preuves pour assurer l'ancrage territorial de l'alimentation. La parole

la crise sanitaire que nous traversons fait cruellement apparaître les conséquences de la délocalisation de certaines productions et de la dépendance croissante de l'Europe à l'égard de chaînes de valeur stratégiques cruciales qu'elle ne maîtrise plus. Les évolutions du secteur du médicament sont à cet égard particulièrement préoccupantes. En effet, 80 % des principes actifs pharmaceutiques utilisés en Europe sont désormais fabriqués hors de l'espace économique européen, une grande partie en Asie, plus particulièrement en Chine et en Inde. Dès lors, il suffit d'une catastrophe naturelle ou sanitaire, d'un événement géopolitique ou d'un accident industriel pour entraîner des ruptures d'approvisionnement pouvant conduire à priver les patients européens des traitements indispensables. Incontestablement, la maîtrise de la fabrication des matières premières à usage pharmaceutique apparaît aujourd'hui comme un enjeu stratégique national et européen, tout comme la synthèse des substances actives, voire de certains excipients indispensables à la formulation La stratégie pharmaceutique sur laquelle travaille la Commission européenne s'inscrit dans cette logique de relocalisation en Europe des antibiotiques ou des anticancéreux. Elle devra s'assurer de la disponibilité, du caractère abordable, de la durabilité et de la sécurité de l'approvisionnement en la matière. La situation de dépendance de notre pays et de nos voisins que la crise sanitaire a mise en lumière n'est pas nouvelle, mais elle s'est accrue au cours des années récentes. Elle est loin, en outre, de ne concerner que le secteur de la santé. Il est donc urgent de réagir et de s'assurer que l'Europe est en mesure de maîtriser

de souligner les notions de réciprocité de l'ouverture des marchés, de concurrence équitable et de taxation équitable, au travers des productions décarbonées, sur lesquelles nos entreprises font de gros efforts, ce qui n'est pas le cas, loin de là, dans d'autres parties du monde. La question clé qui est au coeur de notre débat cette après-midi est celle de la détermination des productions stratégiques pour la souveraineté économique européenne. Avant d'agir, il est en effet essentiel de procéder à une analyse fine des secteurs identifiés comme stratégiques. J'avoue que nous ne pouvons que nous réjouir de la détermination et de l'engagement de notre commissaire européen Thierry Breton,

Deux dysfonctionnements majeurs affectent aujourd'hui l'accès aux médicaments : l'accroissement des pénuries de médicaments et, bien entendu, notre dépendance à l'égard de la Chine et de l'Inde. Ces deux dysfonctionnements conduisent à nous interroger sur un troisième,

D'un certain point de vue, l'industrie pharmaceutique est sans doute l'industrie la plus subventionnée dans notre pays. Le rapport entre les dépenses de la sécurité sociale et l'industrie du médicament nous conduit à réfléchir sur ce que devrait être une politique publique du médicament.

Il ne reste plus qu'une centaine de sites de production dans notre pays. Dans le domaine de la production de médicaments innovants, le bilan n'est pas meilleur. Sur 254 nouveaux médicaments autorisés entre 2016 et 2018, seulement 20 sont fabriqués en France. Et le retard est encore plus considérable pour la production de médicaments biologiques.

portée à la connaissance de tous par neuf grands hôpitaux européens en pleine pandémie ! Au quotidien, en 2019, quelque 1 450 médicaments étaient en rupture, dont 14 vaccins.

ce qui permet la réalisation de fortes marges. L'argument de la recherche, souvent avancé, n'est pas totalement honnête. En effet, les résultats en termes de recherche ne sont pas à la hauteur de l'argent public investi dans l'industrie pharmaceutique. La sécurité sociale finance la recherche privée

Le Gouvernement dit aujourd'hui vouloir redresser la barre en repensant notre modèle économique et en assurant la pérennité de notre maillage industriel. Le ministre de l'économie et des finances plaide même pour une relocalisation de l'industrie automobile française.

Lorsque le site belfortain de General Electric, en pleine épidémie de Covid-19, a demandé à ses 240 sous-traitants de réduire de 20 % leur prix à partir du 1 mai, sous peine de ne plus être considérés comme des partenaires de l'entreprise, un rappel à l'ordre de l'État aurait peut-être été salutaire. salutaire. Lorsque la direction de General Electric, deux jours après le déconfinement, a convoqué à Belfort un comité social et économique pour annoncer aux représentants du personnel un programme de délocalisation de l'ingénierie, des activités commerciales, de maintenance et de réparation des turbines, une réaction de l'État n'aurait-elle pas été souhaitable ?

L'exécutif clame haut et fort sa volonté de sauver l'appareil productif français. Qu'attend-il pour intervenir et rappeler ses engagements à la direction de General Electric ? La seconde preuve qui qui témoignerait de la volonté de changement du Gouvernement pourrait se situer sur le terrain du pragmatisme. Comme bon nombre de mes collègues, j'ai été sollicité dès le début de la crise par des entreprises et des bénévoles, tous démunis face à la complexité de notre réglementation.

Les normes et les lourdeurs de la technostructure ne doivent pas provoquer plus de dégâts que le Covid-19. Dans ce cas précis, le remède est simple : un peu de pragmatisme et beaucoup de bon sens. Si j'évoque ces quelques exemples, c'est pour demander au Gouvernement de mieux nous défendre en simplifiant les normes et en les faisant respecter aux industriels étrangers, en formant les jeunes aux métiers de l'industrie et en valorisant ces métiers importants, en développant les politiques publiques territoriales en faveur de l'industrie, en favorisant une meilleure diversification des processus productifs, enfin, en renouvelant la vision stratégique et prospective des pouvoirs publics, cela a été dit par ma collègue. Cela pourrait se traduire par la nomination- enfin ! -d'un ministre de l'industrie de plein exercice, qui s'appuierait sur une direction d'administration centrale dédiée.

Je partage également votre intérêt pour la 5G et la voiture autonome, sujets que plusieurs d'entre vous ont évoqués. Dans son programme, le commissaire Breton pointe un certain nombre de technologies clés. Nous l'avons fait aussi dans le cadre du pacte productif. Benoît Potier a

à produire. Voilà la réalité ! Nous recherchons des investisseurs et des repreneurs et c'est un dossier que suit la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises. Sans l'intervention du ministère de l'économie et des finances, Famar aurait fermé l'année dernière. Je me permets de le rappeler.

permettant de réimplanter des activités de santé en France. Je puis d'ores et déjà vous dire que, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous enverrons des signaux forts dans cette direction. Et puisque vous évoquez les 34 plans industriels, je vous renvoie aux 18 contrats stratégiques de filière, qui sont vivants, bien vivants, et qui avancent.

heure - Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat et d'un vote sur cette déclaration, en application de l'article 50-1 de la Constitution, relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19 Temps attribué aux orateurs des